toutes les violences à l'égard des forces de l'ordre qui ont émaillé certaines des manifestations des « gilets jaunes » depuis le mois de novembre. La condamnation de ces agissements ne saurait cependant occulter le grand nombre de manifestants blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense, ou LBD.

Depuis 2009, le LBD 40 a remplacé le Flash-Ball Super-Pro dans les opérations de maintien de l'ordre, car plus puissant et plus précis. En théorie, son usage est très encadré. Le tireur doit viser « de façon privilégiée le torse, ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs », mais en aucun cas la tête. Pour rappel, en termes de maintien de l'ordre, la France fait figure d'exception. Elle est le seul pays européen à utiliser des grenades explosives l'un des rares, avec la Grèce, l'Espagne et la Pologne, à faire usage des LBD. Votre ministère a lancé le 23 décembre 2018 un appel d'offres pour l'acquisition de 1 280 nouveaux LBD.

de l'insuffisance de la formation à la doctrine d'emploi de ces armes par les forces de l'ordre et de l'efficacité contestée du dispositif de caméras piétons pour encadrer compte-t-il suivre l'avis du Défenseur des droits en interdisant l'usage de ces armes ? La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le

Chaque samedi, nous assistons aux mêmes scènes : un certain nombre d'individus très violents, des casseurs, se mêlent aux manifestations et les font dégénérer, parfois dès le début, plus souvent à la fin. C'était encore le cas samedi dernier sur la place de la Bastille. Ce sont des casseurs extrêmement violents,

La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole, et son peuple crève de faim. Le dictateur de Caracas emprisonne et assassine : 100 morts ces jours derniers, 600 prisonniers politiques régulièrement torturés, 3 millions de réfugiés, plus de médicaments. En revanche, pour la drogue, pas de problème : le plus grand cartel de narcotrafic du monde est supervisé par les militaires vénézuéliens eux-mêmes Deux hommes se prétendent aujourd'hui président de la République : le castro-chaviste Maduro, arrivé au pouvoir à l'issue d'une élection truquée dénoncée dans le monde entier, et Juan Guaido, élu, lui, démocratiquement président de l'Assemblée nationale. Maduro- cela n'étonnera personne -est soutenu par les pays ultra-démocratiques que sont la Russie, la Chine, la Turquie, Cuba, l'Iran et la Corée du Nord. Il est aussi soutenu à fond, chez nous, par le de la France soumise à Cuba, qui repère les dictateurs qui repère les dictateurs avec un flair infaillible : le tyranophile Mélenchon, qui dénonce les violences policières à Paris, mais supporte sans trop de douleur les centaines de morts à Caracas Guaido est reconnu par la quasi-totalité des pays d'Amérique latine et, au total, par une vingtaine de pays du monde. L'Union européenne, qui penche pour Guaido, s'est contentée d'appeler, par ce qu'elle nomme un « ultimatum », à de nouvelles élections.

Trois journalistes espagnols et deux journalistes français ont été arrêtés hier à Caracas. On est sans nouvelles d'eux. L'Espagne a exigé publiquement la libération immédiate de ses journalistes. journalistes. Monsieur le Premier ministre, la France et l'Union européenne vont-elles reconnaître le président Guaido avant qu'il ne soit trop tard et que la guerre civile n'éclate au Venezuela ? Le Gouvernement compte-t-il exiger publiquement la libération immédiate des journalistes français ? Avez-vous de leurs nouvelles ? La parole

Son économie est totalement exsangue, sa population est privée de médicaments et de l'ensemble des biens de première nécessité. Nous parlons d'un pays qui a mis en place une répression sanglante de ses oppositions.

en vue, a-t-il affirmé, d'organiser des élections véritablement démocratiques. Notre responsabilité, celle de la France et celle de l'Union européenne, est de veiller au respect de la volonté du peuple vénézuélien.

est politique, négociée et pacifique. Il y faudra la coopération des organisations régionales et des pays voisins du Venezuela. ministre de l'Europe et des affaires étrangères, est aujourd'hui même à Bucarest avec ses homologues européens pour consolider et affirmer cette position commune face à la crise. La situation humanitaire est préoccupante.

Nous constatons que les délais de jugement ne cessent de s'allonger. Les peines sont mal exécutées. Les prisons sont saturées. Une réforme a été engagée pour répondre à ces difficultés. Cette réforme a suscité une hostilité sans précédent de toutes les professions de justice. Nous avons réuni hier leurs

Il demande au Gouvernement de bien vouloir suspendre les travaux parlementaires pour trouver un accord permettant de faire en sorte qu'une réponse appropriée, pertinente et consensuelle soit apportée aux préoccupations du monde de la justice, que partagent nos collectivités.

Au cours des débats parlementaires qui se sont tenus depuis le mois d'octobre dernier, on a pu observer des points de convergence réelle autour d'un objectif commun : donner enfin à la justice les moyens auxquels elle peut prétendre et la réformer pour prendre en compte les besoins des justiciables.

Votre assemblée est partie d'une position qu'elle avait élaborée dès le printemps 2017 et qui ne correspondait pas aux choix opérés par le Gouvernement après la consultation organisée dans le cadre des chantiers de la justice.

Monsieur le ministre, je regrette de devoir vous dire que cet esprit est un esprit de fermeture. On ne peut pas avoir raison seul contre tout le monde ; on ne peut pas réformer la société par voie d'autorité.

de justice. Le Gouvernement serait bien inspiré, après les troubles des derniers mois, de commencer à comprendre qu'adopter une autre méthode est préférable si l'on veut réformer la société en profondeur. Il faut d'abord rechercher, par le dialogue, davantage de consensus : c'est ce que nous vous offrons de faire

vous avez prévu de réduire encore les services de la direction générale des finances publiques pour faire des économies. On ne peut vous en vouloir, mais ces économies porteront, une fois de plus, sur les territoires plutôt que sur Bercy. Cependant, dans une note préparatoire de décembre 2018, vos services prônaient la concertation locale, la recherche d'un équilibre territorial ou encore l'utilisation de nouveaux outils, comme la téléconférence. Alors chiche, monsieur le secrétaire d'État : osez la concertation, la vraie, car un courrier d'information envoyé à un élu un mois avant l'arrêt d'un service public, ce n'est pas une concertation

il faudrait que les administrations acceptent de collaborer avec ces maisons, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas aujourd'hui. Monsieur le secrétaire d'État, vous qui avez défendu une loi prônant la confiance, comment pensez-vous instaurer confiance et partenariat entre les services publics de l'État et ceux des collectivités locales, afin que tous nos concitoyens aient le même accès au droit ?

vous posez la question de la permanence sur le territoire du réseau de la DGFiP, dont vous avez raison de souligner l'importance. Aujourd'hui, la DGFiP compte 3 800 points de contact, soit un millier de moins qu'il y a dix ans, ce qui témoigne des réorganisations successives. Ces réorganisations, qui se sont traduites par des fermetures, ont un défaut principal : au-delà de la justification de certaines du fait des évolutions technologiques, elles s'inscrivent dans des plans annuels sans visibilité ni pour les agents ni pour les élus locaux. Nous avons demandé, avec Gérald Darmanin, à l'ensemble des services du ministère de l'action et des comptes publics de changer de méthode.

leur demandons d'avoir une vision pluriannuelle de la réorganisation des services de la DGFiP, de manière à donner de la lisibilité aux territoires, aux élus locaux, aux agents et aux contribuables. En deuxième lieu, nous leur demandons de réfléchir à l'échelle des bassins de vie et des bassins d'emplois, en s'extrayant des logiques purement administratives et en travaillant plutôt à l'échelle d'une région, sans tenir compte des frontières administratives du département, bien souvent artificielles au regard du quotidien de nos concitoyens. En troisième lieu, nous leur demandons de veiller à augmenter le nombre de points de contact sur le territoire par tous les moyens possibles le maintien de perceptions, mais aussi le développement de maisons de services au public. Ma collègue Jacqueline Gourault travaille à harmoniser l'offre de services dans les maisons de services au public en veillant à ce que l'ensemble des services de l'État

Les orientations données au ministère de l'action et des comptes publics sont parfaitement conformes aux instructions adressées par le Premier ministre à l'ensemble des ministres pour ce qui concerne la réorganisation des services de l'État sur le territoire.

En 2018, 691 000 nouvelles sociétés ont vu le jour ; le chômage a reculé de 1,5 % en un an le nombre de procédures prudhommales a chuté de 17,61 trois résultats encourageants directement liés à la mise en oeuvre des ordonnances réformant le code du travail et aux actions menées durant ces dix-huit derniers mois. Ces mesures ont permis aux entreprises de se stabiliser, de reconstituer leurs marges et de redevenir compétitives. Leur capacité de sauvegarder, de créer des emplois et de réinvestir s'est renforcée. Nous le savons tous, c'est l'entreprise qui génère la richesse, qui crée de l'emploi et permet à tous de mieux vivre.

Madame la ministre, vous avez lancé, en novembre, la négociation entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage. L'un des objectifs est de lutter contre la précarité, d'inciter les chômeurs à retourner plus vite sur le marché du travail. Or, lundi, les organisations patronales ont décidé de se retirer des négociations, à la suite des déclarations du Président de la République sur le bonus-malus, dispositif consistant à moduler les cotisations chômage de l'employeur en fonction du taux de ruptures de contrats de travail. Cette promesse présidentielle a trouvé le soutien des syndicats, et pour cause : en vingt ans, le nombre de CDD de moins d'un mois a été multiplié par 2,5 Madame la ministre, nous devons continuer à libérer l'économie française tout en protégeant le salarié, et cela ne peut se faire qu'avec la collaboration du Medef, de la Confédération

Casil Europe de la revente des 49,9 % de parts qu'il détient depuis 2015. Les acteurs locaux sont las de ce mauvais scénario, sur lequel je me suis maintes fois exprimée ici. Nous parlons du cinquième aéroport régional et premier aéroport régional de fret, outil de développement essentiel pour le territoire, infrastructure hautement stratégique, notamment pour Airbus, qui en est un utilisateur privilégié. Depuis l'arrivée de Casil Europe, un bras de fer s'est engagé concernant la redistribution des dividendes, l'investisseur privé réclamant « un retour sur investissement raisonnable ». Les collectivités locales n'ont cessé de s'opposer à une politique de redistribution croissante, laquelle a atteint, fin 2018, 100 % des bénéfices Elles n'ont pas été aidées par l'Agence des participations de l'État, qui a systématiquement validé les demandes de l'investisseur privé. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que les derniers 10,1 % des parts appartenant encore à l'État seront bien désolidarisés de la vente par Casil Europe tout nouvel acteur privé ? Je propose d'étudier une vente des parts de l'État aux collectivités locales, qui détiennent déjà ensemble 40 % du capital, afin d'assurer une majorité stable et sereine dans la gouvernance de cet équipement. La parole

en avril 2015, nous avons vendu 49,9 % des parts de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Nous avons mené cette opération dans le respect des règles de droit,

celle de venir me voir avec les autres élus

Sous la pression de l'opinion, vous en convenez désormais et promettez de taxer les GAFAM. Que de temps et d'argent perdus ! Cependant, cette taxation ne doit pas être symbolique. D'abord, le cadre doit être durable. Ces entreprises doivent être taxées comme toutes celles qui sont installées sur notre territoire. Proposerez-vous, comme le Sénat,

Initialement, la France pouvait escompter 1 milliard d'euros de recettes en rythme de croisière. Avec l'accord franco-allemand que vous avez approuvé, ces recettes ne seraient plus que de 400 millions

Il est indispensable de taxer sans délai les géants du numérique. C'est une question de justice personne ne peut accepter que ces multinationales, qui font les profits les plus élevés, payent quatorze points d'impôt de moins que n'importe quelle PME de France ou d'Europe. aussi une question d'efficacité : si nous voulons, demain, pouvoir financer nos services publics, nos crèches, nos hôpitaux, nos écoles, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve ! C'est ce que nous allons faire ! C'est ce que nous allons faire ! À la demande du Premier ministre, nous déposerons dans les prochains jours un projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Cette taxation nationale des géants du numérique touchera toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires numérique est supérieur à 750 millions d'euros et le chiffre d'affaires national supérieur à 25 millions d'euros. La taxation sera progressive, pour que les petits payent moins que les gros

la diffusion d'un documentaire-choc sur France 3, la mobilisation des députés et des sénateurs de tous les bords politiques et l'émotion des Français pour que le Gouvernement se décide enfin à réagir.

Cette confiance, il est de votre devoir de la retrouver. Cette situation dramatique ne date pas d'hier. Les départements, confrontés à la baisse des dotations, à l'augmentation du nombre des placements et des suivis, ne peuvent plus gérer seuls la prise en charge de ces enfants.

Sorties sèches de l'ASE à 18 ans, vieillissement des familles d'accueil, absence de fichier national pour l'agrément : notre système de protection de l'enfance est aujourd'hui à bout de souffle. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, préciser quel est le périmètre de vos attributions et quels seront les moyens attribués à la protection de l'enfance, sachant que rien n'était prévu dans le budget pour 2019 ? En tant que député, vous avez signé la proposition de loi visant à éviter les sorties sèches des jeunes majeurs. En tant que secrétaire d'État, allez-vous soutenir les initiatives parlementaires ?

Je serai le ministre de la concertation et du dialogue franc et sincère, où l'on se dit les choses dans les yeux et où chacun assume ses responsabilités, un dialogue qui associera votre assemblée,

s'adresse à M. le ministre chargé de la ville et du logement, que je remercie de sa présence. Monsieur le ministre, voilà presque deux ans que vous avez pris les rênes de ce ministère, sous une forme ou sous une autre, et les choix du Gouvernement ont désormais des conséquences sur la marche du pays. Force est de constater que la relance du logement a été l'une de vos premières préoccupations. Malheureusement, ce secteur fut aussi la cible des foudres de Bercy. La construction de logements connaît aujourd'hui un sérieux ralentissement. Les chiffres de 2018 sont inquiétants. Le nombre de mises en chantier a baissé de 18 % en 2018,

a atteint, en fin d'année, 27,3 %. Le Gouvernement entendait être jugé sur ses résultats : nous y sommes ! L'exclusion de certaines zones du dispositif Pinel, la fin de l'APL accession, la limitation du prêt à taux zéro, les coupes dans les ressources des bailleurs sociaux,

Madame la sénatrice

Elle a peu à peu progressé vers l'ouest du continent, pour atteindre la Belgique le 13 septembre dernier. Neuf pays de l'Union européenne sont déjà concernés. Deux nouveaux cas ont été détectés en Belgique le 14 janvier dernier, à moins de deux kilomètres de la frontière Non transmissible à l'homme- il faut le rappeler -, la maladie se révèle toutefois extrêmement contagieuse pour les porcins et les sangliers. Les risques d'une entrée en France du virus sont considérables,

L'industrie agroalimentaire ne serait sans doute pas épargnée non plus. Par ailleurs, un fort risque pèse également sur la biodiversité, l'activité forestière et l'économie cynégétique. Vous avez pris des mesures de prévention, monsieur le ministre, dont la mise en place d'une zone blanche où sont éradiqués tous les sangliers, principaux vecteurs de la propagation de la maladie. Je tiens d'ailleurs à saluer la forte mobilisation des chasseurs.

Voilà un an, je l'interrogeais déjà sur les projets de fermeture de classes dans les communes rurales de notre pays. Aujourd'hui, la situation est encore pire : les promesses se sont envolées, des dizaines de classes vont encore fermer et la « France périphérique » se sent plus que jamais abandonnée. En Seine-et-Marne, on annonce près de 180 fermetures, touchant plus de 150 communes sur 507, contre moins d'un tiers d'ouvertures ! Les habitants sont exaspérés, les élus locaux désespérés. Nos villes et nos villages ne pourront pas faire face.

Comment voulez-vous que les maires fassent ? Vous nous parlez chiffres, choix, perspectives, efforts, mais qui fait les efforts ? Nous vous parlons d'enfants qui sont nos adultes de demain et dont le seul tort est de vivre à la campagne, d'équipes d'enseignants qui font un travail remarquable et qui ont besoin de stabilité, de villes et de villages dont le dynamisme va être anéanti, de territoires qui souffrent et que vous refusez d'entendre ! Après les entreprises, les commerces et les médecins, ce sont maintenant les écoles

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Ces dernières années, de nombreux Français ont rejoint les rangs de l'État islamique au Levant. Acquis à la cause salafiste, portés par la volonté de contribuer au djihad armé, ils se sont rendus tristement célèbres par leurs exactions exactions contre les populations locales pour imposer l'ordre tyrannique de Daech. Ils voulaient aussi mettre la France à genoux. Certains d'entre eux, utilisant les réseaux sociaux, ont largement diffusé leur propagande visant à encourager de jeunes Français à les rejoindre ou à commettre des attentats sur notre sol par tous les moyens. Aujourd'hui, un certain nombre de ces individus dangereux, capturés en Syrie, sont détenus par les forces kurdes. Le désengagement américain du Levant pose la question du devenir de ces prisonniers, qui pourraient revenir en France. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il protéger efficacement les Français de ces criminels, de ces ennemis de la République, alors que la menace terroriste reste très élevée dans notre pays ?

C'est pour garantir la sécurité des Français qu'un certain nombre d'opérations ont été conduites contre des terroristes qui, quelle que soit la nationalité dont ils pouvaient se prévaloir, étaient des ennemis. Ils ont été traités comme tels.

eu des enfants. Certains ont été tués dans les combats, d'autres sont aujourd'hui détenus par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie.

Kurdes. Or la décision unilatérale des États-Unis de se désengager de Syrie a suscité chez les Kurdes des interrogations considérables.

Monsieur le Premier ministre, il faut dire la vérité aux Français. Ces prisonniers seront-ils échangés par les milices contre des prisonniers kurdes détenus par Daech ? C'est un risque que vous n'avez pas évoqué. Par ailleurs, la réponse judiciaire envers les « revenants » majeurs est, vous le savez, tributaire de la preuve. Ils tenteront tout pour minimiser leur rôle. Un dossier judiciaire fragile, c'est l'assurance d'une condamnation faible et d'un retour dans la société à brève échéance. Cela n'est pas acceptable. Enfin, c'est un problème dont l'Europe doit se saisir, car les djihadistes comptent de nombreux Européens dans leurs rangs. La charte de Londres et le statut de Rome, vous le savez, le permettent. Nous parlons ici de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Je crois que votre volte-face n'est que le marqueur d'une certaine faiblesse de notre politique étrangère au Levant. Ces personnes ne doivent pas revenir.

d'autonomie qui ont été adoptées par la commission spéciale. Il revient notamment sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d'autonomie. En effet, cette disposition pourrait créer une incertitude sur la période de liquidation de la rente de nature à renchérir la tarification. En contrepartie, l'amendement prévoit l'introduction d'une garantie complémentaire au contrat, visant à prévenir les risques liés à la perte d'autonomie du titulaire.

Cette interdiction, introduite en commission, n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les entreprises ni avec les partenaires sociaux et soulève un certain nombre de difficultés.

C'est pourquoi il serait pertinent que les salariés soient accompagnés et informés à tout moment, notamment lorsqu'ils optent pour la liquidation de tout ou partie de leurs droits par l'acquisition d'une rente viagère à l'ouverture du plan. la mise en place du plan d'épargne retraite, est prévue la transférabilité entre les produits d'épargne retraite existants. Ainsi, il serait possible de transférer à tout moment des avoirs placés sur un support collectif, tel le PERCO, vers un support individuel,

La commission spéciale du Sénat est allée plus loin, en adoptant un amendement visant à abaisser ce taux à 10 %. Notre amendement a pour objet de supprimer ces dispositions, afin de maintenir le taux actuel Pour rappel, le forfait social est une contribution versée par les employeurs qui sert à financer la sécurité sociale. Supprimer ou réduire le taux du forfait social revient à priver notre système de solidarité nationale de ressources pourtant nécessaires à son fonctionnement.

a pu indiquer après avoir été interpellée par notre groupe à la suite de l'annonce récente de la fermeture de la maternité de Creil. Les mobilisations des personnels de santé, qui dénoncent leurs conditions de travail désastreuses et se trouvent souvent

Pour toutes ces raisons, les entreprises doivent continuer de contribuer au bon fonctionnement de notre système de solidarité. Nous entendons les revendications des petites et moyennes entreprises, qui réclament un allégement de charges, et nous ne les confondons pas avec les grosses entreprises. Pour autant, nous refusons que leur financement passe par la destruction

est à Mme Laurence Cohen. Nous sommes, vous le savez, fortement opposés au recours à la procédure d'habilitation à légiférer par ordonnances. C'est une atteinte aux droits du législateur

en vingt-huit alinéas. Elles concernent les conditions de participation des salariés à la gestion des fonds d'épargne retraite, les conditions de constitution de l'épargne, ses règles de prise en compte au titre de l'impôt sur le revenu, l'adoption de dispositifs éventuels de revalorisation ...

on continue à mentir au grand public sur les « injustices » qui découleraient de la spécificité de certains régimes au regard du régime général. De fait, le champ de la réforme se trouverait réduit, et la fameuse « réforme systémique » lestée dès l'origine par la sophistication des dispositifs d'épargne retraite. Notons d'ailleurs tout de suite que l'affaire de la retraite par capitalisation concerne autant, au travers les 150 euros mensuels des plans d'épargne « Fillon » que les plans à prestations définies et pouvoir d'achat garanti, appelés « retraites chapeau » en français grand public. Nous refusons évidemment cette dichotomie savamment organisée dans le débat sur les retraites et nous ne pouvons qu'appeler le Sénat à se saisir de la question, en

concerne les obligations d'information et de conseil relatives aux produits d'épargne retraite collectifs et individuels. Il vise à proposer un compromis. La rédaction actuelle, issue des un compromis. La rédaction actuelle, issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit que ces obligations s'appliqueront pendant l'intégralité de la durée de vie du produit, c'est-à-dire durant la phase d'épargne et celle de la restitution de l'épargne. Cette rédaction n'est pas tout à fait satisfaisante et elle comporte des risques de lourdeur et d'insécurité juridique. Elle risque aussi de conduire les assureurs

et est susceptible d'engendrer une baisse de la rémunération des contrats tant d'épargne que de retraite. Au contraire, une mutualisation des fonds permet de diversifier les risques et de rendre les actifs peu sensibles aux variations de taux Elle favorise la création de fonds propres qui sont investis sur des actifs d'horizon beaucoup plus long, apportant de ce fait une rémunération complémentaire au bénéfice des épargnants et des futurs retraités. Enfin, elle favorise les investissements en actifs permettant le financement en fonds propres des entreprises françaises.

car si la portabilité des droits contribue à l'attractivité du plan d'épargne retraite, elle ne doit pas se traduire par une déstabilisation d'un outil collectif du dialogue social au sein de l'entreprise.

Sur l'amendement n° 805 de M. Yung, l'avis est favorable, puisqu'il supprime une disposition venant contraindre les possibilités de transfert de plans d'épargne retraite d'entreprise.

la transférabilité, en interdisant le transfert d'un plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise du salarié. Tout ce qui limite la liberté du citoyen sans motif véritablement solide ne me semble pas aller dans la bonne direction. L'avis est donc défavorable.

mais nous sommes là pour défendre l'épargnant plus que l'assureur. Eh oui ! Le cantonnement est une mesure essentielle dans la réforme de l'épargne retraite. Je me permets d'insister sur ce point : supprimer le cantonnement, c'est porter une atteinte directe aux droits et à la protection des épargnants.

Le Sénat a eu à coeur, ces dernières années, et notamment lors de l'élaboration de la loi Eckert de 2014, de renforcer les dispositions protégeant les bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d'être encore renforcé. En particulier, l'information dispensée aux bénéficiaires de contrats d'assurance vie est encore lacunaire. La loi ne prévoit ainsi ni obligation d'informer le bénéficiaire du montant du capital de l'assurance vie à la date du décès de l'assuré et des intérêts produits par ce capital après cette date,

obligation aux assureurs. Mes chers collègues, je vous appelle à adopter ces mesures, qui s'inscrivent dans le prolongement des dispositions adoptées ces dernières années par le Sénat, visant à renforcer la protection des bénéficiaires de contrats d'assurance vie.

Mais tout cela, c'est de l'enfumage

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article vise à rendre nos entreprises « plus innovantes », en permettant d'« améliorer et diversifier les financements », notamment en prenant des mesures « en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés Il s'agit de mobiliser plus ou moins 10 milliards d'euros, issus du produit de la cession d'entreprises publiques stratégiques et du dégel de l'épargne réglementée, pour favoriser l'innovation dite « de rupture n'avons-nous pas déjà quelques outils pour atteindre cet objectif sans recourir à l'abandon des actifs d'État et sans s'attaquer à l'assurance vie ? Que faisons-nous, par exemple, du dispositif Madelin, que nous aurions pu nous contenter de renforcer pour inciter ceux qui en tirent aujourd'hui parti à en faire un peu plus ? Comment justifier une telle mesure quand vous refusez toujours ne serait-ce que le moindre débat sur l'ISF et son rétablissement ? Pourtant, je le disais, cet impôt couplé au dispositif ISF-PME constituait une incitation forte à des investissements dans la production. Sans même parler d'un renforcement de cet impôt par une augmentation de son taux et des contribuables concernés, sans parler d'un élargissement de son assiette, un rétablissement répondrait à l'objectif que vous vous êtes fixé d'augmentation des investissements des particuliers en direction des entreprises. Et tout cela sans compter sur le milliard d'euros mobilisé par l'ISF-PME, un millième du patrimoine global estimé fin 2017, souvent égaré dans les frais de gestion des fonds de « défiscalisation Il ne fallait donc pas grand-chose, monsieur le ministre, pour que le financement de nos entreprises soit porté par des mesures qui sont loin d'être aussi risquées que celles qui sont préconisées. Celles-ci portent, certes, des traces d'une innovation de rupture en matière de gestion des affaires publiques, mais je

Je vous remercie,

Je partage votre volonté de sécuriser l'avenir, de participer à la réussite économique des entreprises, au dynamisme de la France et même au financement de l'économie productive.

! En effet, notre débat est intéressant : derrière la loi PACTE, il y a un débat sur ce que nous voulons pour l'économie française. Je ne cesserai de redire que notre économie a besoin de produire plus, d'investir, d'innover, de créer des emplois et d'avoir du capital à sa disposition. Et je continuerai de dire que les choix fiscaux fiscaux faits par le Gouvernement en 2017, que j'ai présentés ici au Sénat et à l'Assemblée nationale, et qui visaient à diminuer la fiscalité sur le capital en France, sont justes et nécessaires pour notre pays.

! Je ne sors pas de cette logique. Elle est différente de la vôtre, mais je constate, tout simplement, que le chômage a baissé depuis deux ans. Même si ce n'est pas suffisant, nous sommes dans la bonne direction.

Je ne dis pas que tout cela est parfait. Je pense que l'on peut faire beaucoup mieux, car les entreprises françaises ont le talent pour faire beaucoup mieux si nous adoptons des dispositions pour leur faciliter la vie et soutenir l'investissement. Mais je considère que nous sommes dans la bonne direction.

Tout l'objectif de cet article, c'est d'inciter les Français à aller davantage vers ces produits qui financent directement l'économie française. Je veux rassurer M. Gay et l'ensemble des sénateurs, nous aurions pu proposer le « grand soir » de l'assurance vie.

sa philosophie générale me gêne un peu. Au fond, monsieur le ministre, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une épargne passive, qui ne sert pas à grand-chose, tout simplement parce que nos concitoyens ne souhaitent pas prendre des risques.

ce qui fait l'avenir de notre économie, c'est l'investissement à réaliser. Or, lorsque l'on sait que la quasi-totalité ou la majeure partie des bénéfices servent simplement à rémunérer les actionnaires et non pas à financer l'investissement, il me semble que

que nous aurons l'objectivité et la neutralité nécessaires pour leur faire valoir les avantages et les inconvénients des diverses solutions qui existent sur le marché.

à des mécanismes de finance verte encore beaucoup plus efficaces. Ceux-ci reposeraient sur un principe de transparence, grâce auquel on pourrait évaluer très précisément la part d'actifs de chaque banque

Est-elle dirigée vers des énergies renouvelables, vers des centrales ou des mines à charbon ? Je suis convaincu que, au bout du compte, ceux qui feront la finance verte, ce seront les clients.

la transition énergétique plutôt que dans une banque qui continue à financer des activités qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. C'est une conviction très forte chez moi. Toutefois, votre amendement me pose problème pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. En effet, vous touchez au droit des contrats parce que vous remettez en cause des contrats déjà conclus. conclus. Pour l'avenir, nous avons déjà prévu des dispositifs qui permettent d'orienter l'épargne vers l'assurance vie verte, mais nous ne souhaitons pas remettre en cause les contrats déjà conclus. C'est la raison pour

explication de vote. Monsieur le ministre, j'entends bien vos explications. Je crois néanmoins que l'urgence climatique actuelle nous oblige à jeter un regard différent sur cette situation. Alors que les participants aux différentes manifestations pour le climat regroupent un nombre toujours plus important de personnes, il ne nous paraît pas tout à fait incongru de permettre la présentation d'unités de comptes véritablement responsables, puisqu'il s'agit bien d'une simple possibilité qui serait donnée à l'ensemble des contrats.

dans l'épargne de long terme orientée vers la production à partir de produits à risque, à savoir les actions. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, l'assurance appartenait à l'État était sous l'autorité et la tutelle d'une direction des assurances. Les produits vendus aux clients étaient labellisés par l'État. Or, involontairement- c'était avant le numérique, je le reconnais

était de protéger la veuve de Carpentras, de telle sorte qu'elle puisse vendre ses actions dans le cadre de son assurance vie ou de son contrat de capitalisation avec un cours connu. Or, aujourd'hui, avec la réactivité des cours, tout se sait en instantané et même un décalage de deux ou trois jours- ce sont souvent des contrats d'une semaine, voire de quinze jours -, vous donne la certitude de vendre ce qui baisse

et de jouer des sommes considérables, de faire perdre la banque, laquelle va s'équilibrer sur les autres épargnants, créant ainsi un déséquilibre absolu. C'est un problème juridique extrêmement complexe. Je pense que seul le législateur peut intervenir, car les autorités de tutelle qui ont succédé à la direction des assurances ne peuvent intervenir qu'après, quand le mal est constaté. Les dispositions de l'amendement ici s'inspirent d'une idée simple et constitutionnellement acceptée : lorsqu'il y a un risque né d'une mutualisation, il faut le limiter. Nous prévoyons l'indemnisation. Je suis heureux d'ouvrir ce débat, qui ne sera peut-être pas tranché aujourd'hui, mais qui aura au moins le mérite d'être posé.

Je crains que le scandale d'une martingale que nous aurions laissé filer en toute connaissance de cause ne provoque chez les épargnants le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures et des traitements différents. C'est la raison pour laquelle,

dont les encours serviront au financement de la transition énergétique et écologique. Ces contrats se caractériseraient par une prime unique, investie, pour au moins 50 %, en faveur de la transition écologique. Cet investissement se répartirait entre des fonds portant un label contrôlé par l'État. s'engagerait sur le long terme, sans possibilité de rachat pendant une durée de huit ans, mais avec la certitude de pouvoir bénéficier d'avances. Par ailleurs, le contrat bénéficierait d'engagements de l'assureur en matière de conditions financières minimales, notamment en termes de frais de gestion et d'avances. Pour répondre rapidement aux besoins de financement de la transition écologique, chiffrée à près de 40 milliards d'euros par an, et afin de stimuler l'offre des assureurs, les encours actuels pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Pour être pleinement efficaces, afin d'accompagner et de sécuriser les épargnants, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finances d'une garantie de l'État. Ainsi, cet amendement tend à concrétiser l'ambition d'un engagement clair et ferme de la France en faveur de la transition écologique. Il s'agit là d'une véritable sécurité pour une épargne responsable, c'est-à-dire une épargne véritablement au service des générations futures. Quel

Au regard des consultations et des informations que nous avons pu recueillir, la collecte de ces fonds ne s'élève aujourd'hui qu'à environ 4 milliards d'euros, ce qui, vous en conviendrez, est bien peu au regard des encours de l'assurance vie. la commission spéciale a adopté une disposition visant à renforcer l'obligation de proposer d'investir dans des fonds verts, solidaires et responsables, ce qui me semble constituer une première étape.

je dis bien pourrait -constituer un effet d'aubaine important pour des souscripteurs qui se détourneraient rapidement de ce fonds. En effet, on pourrait investir dans un

Enfin, pour avoir eu des contacts avec les promoteurs de ce projet, je suis également réticent au regard des différentes modalités d'une rapidité extrême

Ainsi, on ajoute un nouvel élément, qui va complexifier encore l'assurance vie. Il existe déjà trois types de contrats d'assurance vie ; on en créerait un autre, alors même que l'on a demandé aux assureurs que leurs unités de compte comportent des produits verts.

: cela peut provoquer des comportements complètement irresponsables de la part des assureurs. Sachant qu'ils sont couverts par une garantie d'État, ils peuvent prendre tous les risques qu'ils veulent, en promettant à leurs clients une rentabilité exceptionnelle : si cela marche, tant mieux pour eux ; si cela ne marche pas, c'est le Trésor public qui paiera.

: La parole est à M. Michel Vaspart. Cet amendement vise à compléter le cadre légal, qui prévoit la procédure de versement d'une assurance vie à son bénéficiaire. Lorsque celui-ci a été identifié, la loi prévoit que l'assureur a quinze jours pour lui demander des documents, afin de procéder au paiement ensuite d'un délai d'un mois pour verser la somme. Si ce second délai est subordonné à des pénalités en cas de non-paiement, aucune sanction n'est en revanche prévue en cas de manquement au délai de quinze jours. Or, comme a pu le relever le médiateur de l'assurance, cette absence de pénalité favorise le dépassement de cette échéance prévue par la loi. Des délais de plusieurs mois, au lieu des quinze jours légaux, sont parfois observés. Aussi, il s'agit de soumettre le non-respect de ce délai à des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois, puis au triple du taux légal, sur le même principe que celles qui sont appliquées en cas de manquement au délai d'un mois

Concrètement, pour avoir un impact sur l'épargne des Français de manière à financer l'économie réelle, il faut s'attaquer au stock d'assurance vie. Comme cela a été également rappelé, sur les 1 700 milliards d'euros d'assurance vie, 80 % sont investis dans des fonds euro, soit un capital garanti, mais qui ne finance pas l'économie. des marchés financiers, l'AMF, c'est dû à une offre des banques de réseaux souvent pauvre en supports d'investissements ou à des conseillers bancaires insuffisamment formés au conseil de gestion de patrimoine. 74 % des détenteurs de contrat d'assurance vie aimeraient pouvoir transférer celui-ci comme bon leur semble, de manière à avoir une meilleure gestion et un meilleur service. En effet, les détenteurs de contrat gardent leur épargne sur le long terme, notamment pour préparer leur retraite ou laisser un capital à leur succession. Or la loi n'autorise pas les transferts des contrats d'assurance vie. Un épargnant qui détient une assurance vie et qui souhaite changer d'assureur, de courtier ou de conseiller est obligé de mettre un terme à son contrat et d'en contracter un nouveau.

il perd définitivement les avantages successoraux pour les primes versées et produits attachés avant cet âge. Ce matin, monsieur le ministre, vous avez affirmé qu'il était « de notre responsabilité de proposer des produits plus attractifs ». Cet amendement vise à permettre la transférabilité des contrats d'assurance vie, en prévoyant que le transfert d'un contrat n'emporte pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Il est précisé que le dénouement ne peut avoir lieu qu'au bout de huit ans, soit la durée requise pour l'application du régime fiscal de l'assurance vie, afin de permettre une détention relativement relativement longue des fonds dans un premier outil de portage.

Je vais essayer de tenir en moins de huit minutes,

Lavarde, je propose que nous retravaillions ensemble sur la concurrence entre les produits d'assurance vie. En revanche, la portabilité et la transférabilité des contrats d'assurance vie, telles que vous les proposez dans cet amendement, me paraissent

L'assureur ne pourra pas investir en actions, qui est un placement de long terme, à partir du moment où il sait que l'assuré peut changer de contrats d'assurance vie quand bon lui semble.

nous faut donc faire un choix entre le développement du financement en actions de notre économie, le développement des produits en actions de l'assurance vie et la transférabilité des contrats, qui provoquerait un va-et-vient permanent de la part des assurés. Nous faisons le choix du financement en actions stable et durable pour notre

aux assureurs pour avoir des placements en actions me semble tout à fait excessif par rapport au risque que cela représente. La première raison, c'est donc le des assurés, qui fera baisser la part en actions de l'assurance.

La troisième raison est de principe. La fiscalité des contrats d'assurance vie, à laquelle je n'ai aucune intention de toucher, est extraordinairement favorable. Pourquoi ?

le financement de l'économie. Il vise à garantir un bon financement stable et de long terme de l'économie. Si l'on garantit la même fiscalité attractive, tout en permettant à l'assuré de changer de contrat tous les quatre matins, en fonction du niveau des taux et en fonction de son intérêt, on s'expose à un vrai problème de principe quant à l'avantage fiscal qui est accordé. Pour les trois raisons que je viens d'exposer, je vous propose de En revanche, vous mettez le doigt sur un sujet très juste : aujourd'hui, il n'y a pas assez de concurrence entre les assureurs et entre les différents produits pour permettre plus de transparence,

vie est capté par quelques gros assureurs et banques, dont l'AMF a souligné la relative incapacité à orienter les épargnants vers des sources de financement de l'économie réelle. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre,

des formules pour introduire un peu plus de concurrence dans ces dispositifs, tout simplement parce qu'ils engagent les gens pour de très longues années, parfois des décennies.

pourquoi adopter des dispositions comme celles que vise à introduire cet amendement permettrait d'avancer sur la prise en compte d'objectifs un peu plus ambitieux pour notre pays et donnerait aussi un peu plus de liberté à l'ensemble des épargnants. Il n'est pas normal qu'il y ait des rentes assurées pendant des décennies pour un certain nombre d'opérateurs du marché.

il convient tout de même de ne pas oublier que solliciter les marchés financiers, plutôt que ses ressources propres, revient à s'endetter et à assumer les conséquences d'un choix pour le moins coûteux. veut réformer l'épargne retraite, ce qui nous offre l'article 20, qui cherche à aller plus loin que le cadre fixé en 2003 par la réforme des retraites de François Fillon. Il s'apprête à séparer l'assurance vie de sa fonction essentielle de financement de l'endettement public, pour le conduire vers le placement en actions.

Une compagnie d'assurance vie proposant un produit multisupports pourra toujours prendre dans son portefeuille une partie des émissions obligatoires prévues à l'article 22 ou quelques-unes des actions proposées à la vente. Le chemin emprunté est le même que celui qu'ont pris les États-Unis il y a quelques années, avec une réussite économique et sociale largement discutée et discutable. Dans un contexte économique où le taux directeur de la Banque centrale européenne demeure fixé à zéro, et où celui qui frappe les excédents est maintenu à 0,4 %, vouloir passer par les marchés financiers s'apparente, selon nous,

Le CAC 40 représente, pour cette année, près de 47 milliards d'euros de dividendes, sans compter environ 11 milliards d'euros en rachats d'actions, pour une capitalisation boursière de 1 400 milliards d'euros, c'est-à-dire une

soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes, sans que cela ait d'impact véritablement positif pour l'économie. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement préconisent la suppression

les contraintes réglementaires, notamment les obligations de transparence imposées aux entreprises cotées ; enfin, le fait qu'une introduction en bourse ne soit plus le but ultime des entrepreneurs. d'adopter cet article, il me semble que le Gouvernement passe outre ce dernier élément et tente quelque peu de tordre le bras des entrepreneurs. Pourtant, je pense qu'il y a dans les réticences des entreprises un fond de bon sens, d'autant d'autant que, si la baisse des cotations a démarré peu ou prou en même temps que la crise des, ce n'est certainement pas une coïncidence. Peut-être aurait-il été préférable que le Gouvernement tende un peu plus l'oreille vers les dirigeants d'entreprises et, notamment, de PME, car ces derniers ont compris certaines choses.

la bourse, des coûts inhérents à toute cotation, au travers des prix d'entrée et de maintien, mais aussi de toutes les dépenses annexes, notamment pour le conseil et le suivi boursiers. Ils n'ignorent pas, deuxièmement, que les structures les plus à même d'accompagner les entreprises dans leur développement, notamment en matière d'investissement, sont les banques, de mener des opérations d'endettement contrôlé. Il s'agit ici de rappeler la responsabilité des établissements bancaires en matière de participation à l'économie réelle,

a fait le choix du plus élevé, qui s'élève à 8 millions d'euros. De fait, on peut s'interroger sur les raisons qui pousseraient des investisseurs à s'engager dans un projet alors que l'entreprise demandeuse ne fournit pas un bilan de sa santé et de sa situation. Nous avons donc un doute

nous pouvons comprendre la nécessité d'une ordonnance pour simplifier, dans leur lisibilité, le code de commerce et le code monétaire et financier. Cette démarche fait l'objet suite aux recommandations formulées par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris dans son rapport portant proposition en vue de la création d'un chapitre du code de commerce dédié aux sociétés cotées. nous sommes beaucoup plus réservés, voire hostiles, quant aux demandes d'habilitation relatives au régime des offres publiques de titres financiers et, surtout, à la réforme du démarchage bancaire ou financier. Ce démarchage est défini par le code monétaire et financier comme toute toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d'opérations sur une série d'instruments financiers fourniture d'un service d'investissement ou d'une prestation de conseil en investissement ; la liste n'est pas exhaustive ! Le démarchage recouvre encore « le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins nous débattons vise à conforter le financement participatif, voire à lever l'interdiction du démarchage bancaire et financier pour certains instruments financiers non cotés. Le Gouvernement cherche à mettre le droit français en conformité avec le droit européen, mais en abaissant la protection de nos concitoyens

de produits titrisés, dérivés et hybrides, et par d'autres montages malheureux ruinant l'épargne péniblement accumulée par ces ménages que vous avez défendus, monsieur le ministre ? Nous estimons quant à nous que ces thématiques sont trop importantes pour ne pas être discutées pleinement par la représentation nationale, d'où notre demande de suppression de ces alinéas.

responsables d'abus de majorité ou de minorité. En effet, il n'existe pas aujourd'hui en France de dispositif juridique protégeant efficacement les PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.

L'intégration dans la loi d'un tel droit de retrait et d'un droit d'exclusion des actionnaires minoritaires se justifie par le caractère insuffisant de l'indemnisation actuellement octroyée lors de conflits entre actionnaires.

On se retrouve ainsi dans des situations qui sont nuisibles à la vie des entreprises. Il faut donc essayer d'y remédier : tel est l'objet de ces amendements, qui sont dans le droit fil du rapport du Haut Comité juridique de la place

Ces dispositifs sont complexes. En outre, ils reposent sur des notions juridiquement incertaines. Dès lors, de mon point de vue, ils nécessitent une réflexion plus approfondie, à la mesure des changements qu'ils représenteraient pour le droit des sociétés. En effet, l'objectif affiché des auteurs de ces amendements est d'inciter des investisseurs à entrer au capital de PME non cotées, tout en restant minoritaires. Le bon outil, dans ce cas de figure, outre des statuts

qu'il a été complété par la commission, il permet notamment de faciliter le retrait du capital. J'estime qu'il faut prendre garde, en droit des sociétés, à ne pas procéder à des ajustements à résoudre des problèmes particuliers, posent de véritables incertitudes constitutionnelles relatives au droit de propriété.

permet donc, dans la plupart des cas, de résoudre ces difficultés.

puisque l'article 23 constitue, de fait, un projet de loi à lui tout seul, qui vise à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris, notamment dans le contexte du Brexit. Depuis la décision britannique, la City est devenue un enjeu pour tous les pays boursiers d'Europe. C'est sur cette base que le Gouvernement est déjà revenu sur les engagements de ses prédécesseurs, notamment en matière de taxation sur les transactions financières en faveur du développement et de la solidarité internationale.

Quand bien même un tel exode aurait lieu, la mise vaut-elle le sacrifice fait et les risques encourus ? Nous ne sommes pas convaincus que le développement de l'industrie financière soit une solution socialement et économiquement acceptable pour notre pays. Si la place financière occupe, dans les raisonnements économiques, une place secondaire, elle s'inscrit toutefois dans l'économie réelle, non pour la développer, mais bien dans une perspective prédatrice de captation de la valeur créée par les entreprises. Les bulles spéculatives et les crises qu'elles engendrent ont montré toutes les limites de ce secteur, et ce bien avant 2008, voire 1929. De fait, on ne peut que douter de l'énergie déployée jusqu'ici par le Gouvernement. Enfin, quand bien même les 20 000 salariés que j'évoquais quitteraient Londres, Paris serait-il leur premier choix ? Il faut rappeler que la capitalisation boursière de l'ensemble des valeurs inscrites à la cote du CAC 40 est aujourd'hui à peine supérieure à celle des deux premières valeurs du Dow Jones. Pour ne prendre que deux exemples, Microsoft et Apple disposent aujourd'hui d'une capitalisation voisine de quelque 1 380 milliards d'euros, comparable donc avec la valeur du CAC

de l'ensemble de l'activité financière mondiale, et ce dans toutes les devises possibles et imaginables, ce qui fait sa force.

au-delà de la modification de certaines règles portant sur les produits dérivés, vous dispensez temporairement d'affiliation au régime obligatoire de retraite les salariés qui seraient relocalisés à l'avenir en France. Vous excluez les bonus récupérables du calcul de l'indemnité de licenciement, ce qui la fait baisser. vous complétez le régime juridique des succursales d'investissement en France et vous élargissez les modes de négociation des titres de créances négociables. Cet article comporte aussi des transformations non négligeables de la structure des marchés financiers, au profit de ces mêmes marchés de la réalisation d'opérations financières qui n'ont pas forcément pour but de financer l'économie. Je relève un seul point positif : le renforcement des pouvoirs de l'AMF de suspendre les marchés en cas d'événement exceptionnel ; ce pouvoir inclut désormais les plateformes autres que les marchés réglementés.

M. Fabien Gay. Ces alinéas créent deux dispositifs qui permettent aux entreprises employant des traders de les sanctionner s'ils effectuent des placements à risque qui entraînent des pertes. D'une part, les entreprises sont ainsi autorisées à récupérer les bonus versés à leurs salariés ; autrement dit, elles peuvent retenir sur le salaire de leurs traders les sommes qui auraient été perdues en raison de mauvais placements financiers. D'autre part, lesdits bonus peuvent être exclus pour le calcul de leur indemnité de licenciement, laquelle consiste en un pourcentage de la rémunération globale, ce qui conduit nécessairement à la réduire. D'un point de vue juridique, ces deux dispositions sont à notre sens une aberration. Elles remettent en cause un principe central du droit du travail, qui est l'interdiction des sanctions pécuniaires. Cette interdiction se justifie par le fait que l'entreprise créée l'activité, en tire les bénéfices et doit en assumer les risques, sans pouvoir les répercuter sur ses salariés. D'un point de vue politique, ces dispositions sont également répréhensibles. Elles servent clairement à valider la décision de justice en faveur de la Société Générale dans l'affaire Kerviel. J'en profite pour rappeler que le P-DG de la Société Générale, interrogé par la commission d'enquête du Sénat, avait nié le rôle des banques dans la fraude fiscale, alors même que le scandale des permettait de démontrer l'implication de cette banque. Sanctionner les traders qui effectuent de mauvais placements financiers, c'est oublier bien rapidement que ce sont les banques qui organisent le système financier, qui créent des failles et les exploitent. Cela revient à faire peser les conséquences du système financier sur ces salariés qui ne sont bien souvent que de simples exécutants, et auxquels on demande de faire des placements toujours plus risqués, car plus rentables. Ces dispositions visent à sanctionner un individu isolé, en oubliant de faire le procès de la finance. C'est pourquoi nous demandons leur suppression. Espagnac. Le fait de calculer les indemnités d'une personne en ne tenant pas compte de la part variable de sa rémunération crée une rupture d'égalité entre les salariés. Si le secteur incriminé est particulier, cette particularité cette particularité ne saurait justifier une telle mesure d'exception. Il s'agit non pas de protéger un secteur d'activité très lucratif, celui des traders, mais d'éviter l'ouverture de brèches dans les protections aux salariés prévues dans le code du travail. Tous les salariés ont droit au même niveau de protection et une telle disposition, aux conséquences financières par ailleurs lourdes pour les intéressés, apparaît complètement excessive. Les auteurs du présent amendement proposent en conséquence la suppression de cette disposition.

! Enfin, pour nous, l'exception ne doit pas devenir la règle. Si nous ouvrons une seule brèche pour les traders, je pense que, demain- je commence à nous connaître toutes et tous -seront

des loups affamés. Ils doivent être traités comme tout le monde. Il est donc juste qu'un mécanisme permette de vérifier qu'ils ont respecté les règles qui leur sont fixées.

de l'entrée en vigueur du Brexit, les établissements qui opèrent depuis le Royaume-Uni ne disposeront plus du passeport financier européen et deviendront des Pour pouvoir continuer à fonctionner et à exécuter leurs contrats, il faut que des équivalences soient mises en place. Ces équivalences sont partiellement prévues par la Commission européenne. Il s'agit de compléter ce dispositif afin de s'assurer que le régime national d'équivalence applicable aux entreprises d'investissement de pays tiers soit en vigueur tant que l'équivalence européenne n'aura pas été mise en place.

finalement, c'est la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers. Je vais vous dire pourquoi nous cela nous interroge.

article 23 contient une disposition de même nature permettant de transmettre des données de l'AMF à FranceAgriMer.

pour présenter l'amendement n° 126. Le présent article rassemble un ensemble de mesures destinées à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris. Il prévoit la mise en place d'une mesure de dispense temporaire d'affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l'avenir en France. Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans, et son octroi serait conditionné au fait de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années et d'être déjà affilié à un régime d'assurance. Les auteurs du présent amendement sont opposés à une telle mesure qui se ferait nécessairement au détriment des salariés. Ils souhaitent donc la suppression de cette disposition.

Les alinéas 71 à 82 de l'article 23 créent une dispense temporaire d'affiliation au régime de retraite pour les cadres et salariés étrangers qui seraient amenés à travailler durablement en France. L'objectif de cette disposition est de répondre à une problématique soulevée par le rapport du Sénat sur la compétitivité des places financières

Le rapport donne un exemple : sur un salaire de 250 000 euros par an, soit environ 18 000 euros net par mois, le montant des prélèvements obligatoires serait neuf fois supérieur en France par rapport à l'Allemagne- on fait souvent ici des comparaisons avec d'autres pays européens, et bien évidemment avec l'Allemagne ... En clair, cette disposition vise à attirer en France les cadres à hauts revenus, plus particulièrement ceux qui viennent du Royaume-Uni, récemment exclus de la Communauté européenne en raison du Brexit. Une fois encore, les prélèvements obligatoires sont traités comme un handicap par le Gouvernement, alors même qu'il s'agit de contributions visant à financer notre système de solidarité nationale ! Notre sécurité sociale, en attendant que vous la transformiez en protection sociale- vous connaissez la différence entre protection et sécurité est en grave déficit de financement. Pourtant, le Gouvernement accumule les mesures qui la privent de ressources nécessaires : transformation du CICE en allégements de cotisations sociales, non-compensation du budget de la sécurité sociale, réduction du forfait social, et j'en passe ... Le Gouvernement, dans le souci de ne pas trop peser sur les finances des banques, fois d'exonérer les traders et les hauts cadres financiers de l'obligation de s'affilier et de cotiser à notre système de solidarité nationale. Franchement, je trouve cocasse que le Gouvernement s'inquiète du sort de ces traders et hauts cadres financiers,

mesure constitue en effet une réponse bienvenue au principal handicap concurrentiel de la place de Paris, qui a été mis en évidence, je le rappelle- vous l'avez évoqué, mais nous n'en tirons pas les mêmes conclusions -, par la commission des finances du Sénat dans son rapport sur la compétitivité des places financières

et l'activité boursière et financière, l'AMF constitue l'autorité de contrôle chargée du bon déroulement des opérations, du respect des règles prudentielles, de la protection des investisseurs et d'autres fonctions. Cela posé, elle est apparue dès sa création comme une sorte de structure d'autocontrôle des professionnels de la finance par les professionnels de la finance, ainsi que l'illustre sa composition. Le II de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier décrit par le menu la composition de l'instance. Le collège est composé de seize membres qui sont particulièrement monocolores, car ils sont choisis parmi les professionnels de la finance. Le directeur du Trésor participe aux travaux des commissions de l'AMF, sans voix délibérative, et il ne peut siéger à la commission des sanctions, où le poids des professionnels nommés par le ministère de l'économie est déterminant. Quant aux salariés, ils ne sont représentés que par le biais des salariés actionnaires, pour peu que ceux-ci soient éventuellement organisés en association représentative

au monde du travail par le biais de deux représentants issus de nos syndicats confédérés et représentatifs. Cela ne pourra que renforcer l'approche indépendante du fonctionnement de l'Autorité. Quel

que nous proposons, les FIP, dont la souscription est éligible à la réduction de l'impôt sur le revenu PME, devront investir au moins 70 % de leur actif dans une zone géographique constituée d'au plus quatre régions limitrophes. En outre, le fonds ne peut investir plus de 50 % de son actif dans une même région. Afin de renforcer le financement de fonds propres des PME de territoire, il est proposé de réduire cette dernière contrainte à 25 %, ce qui garantira que les FIP investissent dans quatre régions au moins. Cela permettra de diversifier les risques pour les investisseurs et d'élargir l'empreinte géographique des fonds sans supprimer leur ancrage territorial.

Nous n'avons jamais été de fervents partisans-vous le savez -des incitations aux dispositifs défiscalisés ou à fiscalité privilégiée, prétendument destinés à faciliter le lien entre épargne et entreprises. Le dispositif des fonds d'investissement de proximité, les FIP, qui pourrait mériter, comme tant d'autres, une évaluation, connaît surtout un succès d'estime, puisque les derniers chiffres disponibles nous donnent les résultats suivants : une dépense de 23 millions d'euros pour 21 728 ménages dans le cas général, soit un bonus fiscal d'un peu plus de 1 000 euros par foyer fiscal

On sait que, dans les deux derniers cas, le taux de réduction d'impôt est de 38 %, soit environ le double du taux effectif maximal observé en France métropolitaine. C'est donc une dépense de 63 millions d'euros au total qui est imputable à ces FIP,

Cette dépense fiscale est d'un niveau relativement faible au regard des sommes levées, même si elle nous semble quelque peu dépourvue d'un effet de levier significatif. Elle coûte moins cher aux dépenses publiques

peut se faire n'importe où ? Il est donc à craindre que l'instrument ne soit dénaturé et qu'il ne soit utilisé sur la base non pas des besoins de développement local, mais plutôt du seul intérêt du contribuable investisseur à dégager un rendement à partir de l'entourage fiscal de la mesure. Voilà pourquoi nous ne voterons pas cet amendement du Gouvernement.

la création de fonds d'épargne régionaux. Ces fonds permettent aux épargnants d'un territoire donné d'investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui apportera aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont souvent fortement besoin. Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d'investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier, ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d'orientation

par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés dans des PME régionales. Ce dispositif est éligible par nature aux PEA-PME en permettant de rapprocher les épargnants des entreprises de leur territoire. Enfin, une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans cinq régions.

pour le dynamisme économique de nos régions. Cette discussion a émergé au moment de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Nous avons mené plusieurs réunions de travail à Bercy, rassemblant l'ensemble des acteurs concernés issus des différentes régions et plusieurs parlementaires. Ces réunions ont permis d'aboutir à un schéma type de fonds d'investissement régional, qui pourra être mis en oeuvre dans les régions qui le souhaitent, en lien avec les professionnels du secteur financier. Ces travaux ont surtout conduit les participants à la conclusion unanime

L'avantage des FCPR pour les fonds régionaux, c'est qu'ils permettent de s'insérer dans un paysage juridique qui est connu des acteurs, mais également des épargnants. Cela permet aussi de bénéficier du régime fiscal qui existe déjà pour les FCPR et de s'insérer dans des enveloppes de commercialisation, telles

abordons un autre sujet. L'actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d'émetteurs côtés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une fluctuation très pénalisante de leur cours de bourse,

Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter. Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, lorsqu'un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l'intégrité du marché n'est plus assurée. Il confie au président de l'AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d'interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu'à disparition du phénomène.

leurs dispositions entrent en collision- et non en collusion ! -avec le droit européen, qui est venu progressivement, depuis la crise financière, renforcer les dispositifs et encadrer la vente à découvert. en particulier au règlement n° 236/2012 qui prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de restreindre temporairement la vente à découvert d'instruments financiers.

parole est à Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d'une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008. Afin d'empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, l'amendement tend à prévoir une taxation des augmentations de salaires, lorsqu'elles sont attribuées à la fin de la période d'activité des dirigeants de sociétés. Il vise, en outre, la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d'un capital. Il a enfin pour objet de préciser, afin de les limiter, que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net. Quel est l'avis de

dispositif serait difficile à appliquer et paraît risqué sur le plan constitutionnel, compte tenu de la différence de traitement importante qu'il instituerait selon la nature des indemnités versées et leur bénéficiaire.

cet article vise à accroître l'attractivité de la place financière de Paris : il contient des mesures qui assouplissent l'encadrement des infrastructures de marché. Le Brexit se traduira par une mise

assurent la bonne fin des opérations de négociation d'actifs financiers entre les différents acteurs et jouent ainsi un rôle central dans la préservation de la stabilité du système financier. Ce qui pose particulièrement problème à nos yeux, et c'est pourquoi nous avons demandé l'examen de cet article en séance publique, c'est que celui-ci opère une dérégulation de la compensation. Aujourd'hui, seules l'Allemagne et la France imposent systématiquement le statut d'établissement de crédit aux chambres de compensation, mais le projet de sur cette obligation. Cette libéralisation ne nous apparaît pas justifiée, les chambres de compensation étant des acteurs essentiels du système : la surveillance de leurs activités est indispensable pour éviter des catastrophes financières similaires à celles que nous avons récemment connues. En effet, ce sont des institutions qui s'assurent que les obligations de paiement sont bien réalisées et qui, le cas échéant, compensent les acheteurs ayant fait défaut, de manière à amortir le choc et éviter qu'il ne se propage à l'ensemble du système. Or il y a un risque qu'une chambre de compensation n'ayant plus le statut d'établissement de crédit ne soit amenée à prendre des risques inconsidérés,

que la loi doit continuer à obliger les nouvelles chambres de compensation à avoir un agrément. L'argument qui voudrait que les chambres de compensation qui s'établissent en France ne doivent pas supporter de charges administratives et de contraintes supérieures à celles qu'elles auraient à subir dans un autre pays de l'Union européenne ne nous semble pas pertinent au vu des risques

financier en cas de Brexit. La reconnaissance de l'applicabilité des dispositions de la directive Finalité aux systèmes britanniques pour lesquels les établissements français ne disposent pas à ce jour d'alternative apparaît comme clairement indispensable. Quel est

Toutefois, la réponse est-elle aujourd'hui à la hauteur du problème ? Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, car, lorsque l'on regarde le cours de certaines crypto-monnaies, on a de quoi s'inquiéter si un krach Pour ne prendre qu'un seul exemple, un bitcoin vaut aujourd'hui 3 150 euros ; il y a un an, il valait 14 210 euros. Du jour au lendemain, c'est donc toute l'épargne des investisseurs qui pourrait partir en fumée dématérialisée, entraînant dans sa chute une partie importante de l'économie. Au vu des enjeux, faire paraître des codes de conduite et encourager l'AMF à attribuer des labels de qualité aux acteurs vertueux du secteur est, pour notre je le crois, pour l'ensemble de mes collègues ici, une nécessité. De la même manière, créer un régime d'agrément impliquant l'ACPR et interdire aux prestataires n'ayant pas obtenu l'agrément ou le visa optionnel de faire de la publicité en ligne va dans le bon sens. Nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle ce visa est uniquement optionnel. Le Gouvernement justifie sa position en évoquant le libre arbitre des acteurs économiques et en s'appuyant sur le label de qualité attribué par l'AMF. Concrètement, on expérimente en se disant que, avec une bonne communication, les épargnants se dirigeront vers les acteurs ciblés par l'AMF. Quiconque navigue régulièrement sur internet sait que les incitations à l'investissement sont si pressantes et les informations si difficiles à obtenir qu'il y a fort à parier que le tri entre le bon et

plus tard. Votre amendement tend à revenir sur le caractère optionnel du visa délivré par l'AMF pour les levées de fonds en actifs numériques. je me suis moi-même longuement interrogé sur ce caractère optionnel. Il faut toutefois rappeler que les levées de fonds en actifs numériques constituent une forme d'appel à l'épargne publique sur l'ensemble du réseau internet, lequel est par essence transfrontalier. J'ai évoqué précédemment le Luxembourg, qui n'est pas pour vous un paradis, mais qui n'est pas non plus pour moi un enfer : c'est juste le pays voisin et frontalier territoire. Le caractère obligatoire du visa serait très difficile à faire respecter, alors même qu'il risquerait d'envoyer un signal que l'on pourrait qualifier de « contreproductif » aux acteurs désireux de s'établir en France. Un système obligatoire ne pourrait véritablement avoir, me semble-t-il, de portée pratique pratique qu'au niveau européen. Pour cette raison, la commission spéciale a choisi une autre voie, consistant à donner un avantage comparatif très important aux acteurs régulés et à protéger le grand public des offres non soumises au visa. Une mesure interdisant le parrainage, la publicité en ligne et le démarchage pour les offres non régulées a ainsi été adoptée à l'article 26 B du présent projet de loi. Cela répond en très grande partie à l'ensemble de vos préoccupations.

les risques sont nombreux. Par ailleurs, cet amendement tend à renforcer les exigences prévues pour obtenir l'agrément optionnel pour les prestataires de services de conseil, l'obligation préalable de s'enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissements, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement. Il s'agit donc d'une mesure nécessaire à la confiance et à la sécurité financière pour les investisseurs individuels.

Notre souhait, résultant de consignes claires en matière de transposition, était de ne pas aller au-delà de ce qu'imposent les textes européens. Je comprends toutefois que l'amendement adopté par la commission spéciale vise à traduire dans la loi les orientations plus récentes prises en la matière qui datent d'octobre 2018. Si certaines d'entre elles sont déjà claires, comme l'assujettissement des plateformes « crypto » aux contraintes de LCB, d'autres font encore l'objet d'un examen interprétatif au sein du GAFI lui-même.

Pour les autres services, en effet, l'interprétation des recommandations du GAFI est moins évidente, et les risques identifiés par TRACFIN sont pour l'instant de moindre ampleur. Cela justifie de se donner encore un peu temps de réflexion.